menaces et sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer sont parvenues à un accord. Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

En effet, cet amendement émane de nombreux parents inquiets pour leurs enfants qui ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté (JDC) parce qu'ils vivent à l'étranger. Alors que l'organisation de cette journée est obligatoire dans la pratique, la grande majorité des postes diplomatiques et consulaires ne le font pas. Les raisons invoquées sont à la fois d'ordre budgétaire, les postes ne bénéficiant pas d'une ligne budgétaire dédiée, et organisationnelle, faute de personnel suffisant. Surtout, l'organisation d'une telle journée exige la présence d'un attaché de défense, officier habilité à délivrer un certificat de participation. En l'absence de celui-ci, elle ne peut donc être organisée. L'ambassade remet alors une attestation provisoire aux élèves, précisant que cette journée doit être effectuée dans une caserne avant leurs 24 ans, par leurs propres moyens. Or beaucoup auront des difficultés pour remplir cette obligation. Même si l'attestation de report suffit au regard de la réglementation pour l'inscription aux concours et examens d'État, il n'en reste pas moins que les élèves ne sont que provisoirement en règle avec leurs obligations, d'où l'importance pour nos familles de la tenue de la JDC à l'étranger, comme le prévoit la loi. Quel

avec des élus locaux, vise à permettre à l'armée et aux collectivités locales de généraliser au maximum la possibilité pour la population civile d'utiliser certaines infrastructures militaires présentes sur les territoires de la collectivité. Cela peut concerner notamment des piscines ou encore des gymnases. La présence de ces infrastructures au sein de ces communes est une chance pour les habitants. Il apparaît donc opportun qu'ils puissent en profiter pleinement tout en respectant, bien sûr, les conditions d'entraînement des militaires. Le lien Nation-armée n'en sortirait que renforcé.

le ministre.

monsieur le président.

-, vise à souligner l'importance de la montée en compétences des forces armées dans les secteurs mentionnés. Le recrutement d'une réserve opérationnelle plus spécialisée dans ces domaines pallierait les difficultés d'embauches, malgré les nouvelles ambitions de formation pour les armées.

La mise en oeuvre de la sécurité nationale concerne aussi d'autres corps d'État, comme la police, etc. On sort donc du champ de la LPM.

Monsieur Bonneau,

Depuis le protocole de Kyoto de 1997, les Américains ont permis d'exempter les armées de transparence en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Pourtant, un rapport de novembre 2022 du estime que les émissions estime que les émissions de gaz à effet de serre militaires représentent jusqu'à 7 % des émissions de GES mondiales. Ce chiffre est équivalent aux émissions de 85 % de l'ensemble des voitures et supérieur à celles de la Russie. Si les émissions de l'armée française restent opaques, l'ancienne ministre de la défense Florence Parly affirmait en 2019 que c'est parce que ce ministère a l'empreinte environnementale la plus importante de l'État qu'il a l'impérieux devoir d'être un acteur volontaire et engagé de la transition écologique. Les armées consomment chaque année 800 000 mètres cubes de produits pétroliers, dont les trois quarts concernent les avions. L'utilisation de véhicules militaires, d'aéronefs et de navires, y compris lors des exercices militaires, nécessite en effet du carburant, généralement dérivé de combustibles fossiles tels que le diesel, l'essence ou le kérosène. les installations militaires, y compris les bases, les camps et les quartiers généraux, nécessitent de l'énergie pour l'électricité, le chauffage, le refroidissement, l'éclairage. Pour que la France respecte ses engagements climatiques de baisse de 40 % de ses GES par rapport à 1990 d'ici à 2030 conformément à la stratégie nationale bas-carbone, il est indispensable que l'armée française contribue à cet effort et que la LPM intègre cet impératif par l'amendement que nous proposons ici. Quel

Guillaume Gontard. Cet amendement vise à renforcer la coopération en matière de prévention et de résolution non violente des conflits. Le changement climatique a un impact majeur sur les ressources naturelles telles que l'eau et les terres arables. Les sécheresses, les inondations et les variations des régimes de précipitations entraînent des pénuries d'eau et des difficultés d'accès aux ressources alimentaires, ce qui intensifie les luttes entre pays pour le contrôle et l'accès à ces ressources. De même, l'élévation du niveau de la mer, la désertification et la dégradation des terres sont autant de facteurs qui entraînent des déplacements forcés de populations. Ces migrations massives et les mouvements de réfugiés ne cessent d'augmenter, et avec eux les tensions géopolitiques pour la gestion de ces flux migratoires. Les pays riches en combustibles fossiles cherchent à protéger leurs intérêts économiques, tandis que les pays dépendants des importations d'énergie sont vulnérables aux perturbations de l'approvisionnement énergétique. Le changement climatique déstabilise donc États et régions, créant un environnement propice à l'émergence de conflits violents. Il redéfinit les frontières maritimes et terrestres et entraîne ainsi des litiges territoriaux. La gestion durable des ressources, l'adaptation au changement climatique et la coopération internationale sont essentielles pour atténuer les risques de conflits liés au climat. La France doit jouer un rôle actif dans cette démarche et réaffirmer son engagement pour la paix, la sécurité et la stabilité géopolitique. Elle doit être initiatrice en matière de coopération internationale pour la prévention et la résolution non violente de conflits, ce qui passe naturellement par notre politique de développement. J'en profite pour dire ici qu'il est essentiel que le Gouvernement et le Parlement soient aussi scrupuleux pour respecter la trajectoire budgétaire de la loi de programmation relative au développement solidaire que pour celle de la LPM. Quel

en 2019. Il s'agit aider l'AID à irriguer le territoire national et à aller capter l'innovation dans les territoires qui ne seraient pas parisiens, ce qu'elle ne je vous dois quelques explications, mais peut-être m'en devrez-vous aussi quelques-unes. Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous rappeler quelques éléments en vous citant : « Vous m'avez adressé des observations définitives concluant le contrôle mené par la Cour des comptes sur l'opération Sentinelle. La Cour relève en particulier des améliorations apportées au dispositif Sentinelle et sa reconfiguration sur un dispositif opérationnel permanent de 3 000 hommes, un échelon de renforcement programmé à 4 000 hommes

Il s'agit d'une entreprise sensible, étant donné qu'elle est l'un des fournisseurs critiques de Naval Group et qu'elle fournit également la robinetterie dans les bâtiments réacteurs à un quart des centrales nucléaires en service dans le monde. En réalité, la procédure de sauvetage de cette entreprise est loin d'être terminée, puisque c'est la direction du trésor qui a la main sur le contrôle des investissements étrangers. Le chemin semble compliqué. Si l'on en croit la presse, le Gouvernement recherche des fonds français pour racheter Segault. nous demandons à quel moment le Gouvernement sera prêt à engager du capital public. Il conviendrait en effet de garantir des actions et mesures concrètes pour éviter les échecs passés. En tout état de cause, au regard de la répétition des affaires du même type, nous pensons qu'il serait temps que le Gouvernement renforce la législation et la réglementation, afin de garantir la souveraineté nationale sur les industries stratégiques et de défense. Ce renforcement doit passer par des mesures

monsieur le ministre,

au lieu de créer une procédure spécifique aux entreprises de défense. L'objet de l'amendement est de sécuriser la confidentialité de ce recours, compte tenu de la nature particulière de ces entreprises de défense.

de la BITD. Nous souhaitons insister sur l'importance d'une meilleure intégration des industries de défense dans le champ du financement de la Banque européenne d'investissement pour faciliter cette transition aux échelles nationale et européenne.

pour changer de manière radicale la place que nous réservons aux enseignements techniques et professionnels dans notre système éducatif. Cet objectif ne pourra être atteint qu'en engageant un travail de fond pour faire connaître les métiers de l'industrie, et plus précisément de l'industrie de défense. En effet, ces métiers sont toujours présentés de manière stéréotypée. Pourquoi ne pas faire appel au plan France 2030, qui prévoit d'allouer plusieurs millions d'euros au renforcement de l'appareil de formation français pour former jusqu'à 400 000 jeunes demandeurs d'emploi ou salariés par an aux métiers de l'industrie ? Il s'agirait d'allouer une partie de ces crédits au lancement d'une vaste campagne de communication afin de faire connaître et de valoriser ces métiers, non seulement auprès des jeunes en formation initiale, mais aussi auprès des actifs qui peuvent opérer une reconversion professionnelle.

est très longue, et surtout de conserver des compétences essentielles pour la fabrication de matériels très pointus. Avec mon corapporteur Cédric Perrin, nous avons entendu lors de nos multiples auditions les difficultés que les industriels rencontrent pour recruter. En effet, ces métiers ne sont pas suffisamment avons introduit en commission une disposition visant à promouvoir les métiers de l'industrie, notamment auprès des jeunes et des femmes. Par cet amendement, je propose d'associer les industriels à cet effort en les encourageant à participer aux salons étudiants et aux forums sur l'orientation, afin de mieux faire connaître les industries de défense, dont la grande majorité

Les forces spéciales des trois armées auront un rôle clé dans ce contexte et feront l'objet d'un effort pour renforcer leurs capacités d'actions dans des conflits majeurs déclarés ou face à une situation qui constitue une menace pour la Nation et pour contrer les actions hybrides.

il s'agit de préserver son rôle historique de grande puissance maritime et scientifique au niveau mondial. Le rapport pointe la nécessité pour la France de ne pas manquer le tournant des grands fonds marins, comme elle a pu le faire avec les drones.

du littoral français ... Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui se poursuivra, si nous ne freinons pas l'utilisation massive des sonars. Dès les années 1980, les scientifiques ont constaté un lien entre leur utilisation et la mort de cétacés. D'après des études récentes, les sonars militaires à basse et moyenne fréquence peuvent avoir un impact considérable sur une distance de 300 mètres. Or, à cette distance, bon nombre de cétacés ne sont pas détectables. Ayant la capacité d'émettre pendant des heures, ces sonars peuvent causer des répercussions irrévocables sur la faune marine. Les impulsions sonores de ces instruments effraient et désorientent les cétacés et les mènent à la mort. Cette pollution générée par l'utilisation de sonars interfère avec leur faculté à communiquer et à se déplacer. Elle engendre des blessures oculaires, qui, tout en accroissant leur perte de repères, provoquent des changements dans leurs techniques de plongée, d'ordinaire parfaitement calibrées. Et, s'il ne peut plus plonger correctement, l'animal ne peut plus se nourrir. Il est alors condamné à dériver, simplement porté par le courant, en état de malnutrition et de déshydratation, pour aller s'échouer sur une plage. Il ne s'agit pas, avec cet amendement, de contraindre outre mesure notre marine et l'activité de nos sous-marins, mais nous demandons à l'armée de faire tout ce qui est en son pouvoir, sans, bien sûr, compromettre ses missions, pour rationaliser l'utilisation des sonars, afin de protéger au mieux la faune marine, et particulièrement les cétacés. l'avis de la commission ?

pouvant nuire à son bon fonctionnement. De nombreux produits sont utilisés pour accroître la sécurité : c'est ce que l'on appelle « l'antifouling ». À l'heure où, même à faible concentration, les biocides contenus dans les peintures « antifouling » contaminent l'ensemble de la chaîne alimentaire marine, il est temps d'agir plus efficacement. aux prédateurs, en passant par les organismes filtreurs- huîtres, moules, etc. -, aucun animal n'est épargné. Il est également important de rappeler que nous-mêmes, au sommet de la chaîne alimentaire, nous ne sommes pas à l'abri d'en subir les conséquences.

ces produits existent toujours. Nous sommes conscients des efforts que fait la marine nationale pour supprimer les peintures antisalissure, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas encore suffisants. C'est pourquoi nous les encourageons à chercher des solutions alternatives, si possible naturelles.

extrait d'une lettre personnelle adressée par le général de Gaulle à Pierre Messmer le 19 juillet 1962 : « J'ai constaté, notamment dans le domaine militaire, un emploi excessif de la terminologie anglo-saxonne. Je vous serais obligé de donner des instructions pour que les termes étrangers soient proscrits chaque fois qu'un vocable français peut être employé, c'est-à-dire dans tous les cas.

par celle à « l'écosystème des entreprises privées innovantes du domaine spatial » et de supprimer la parenthèse suivante, où est inscrite l'expression « New Space ». On peut comprendre que certaines expressions consacrées, certains concepts internationaux

spatial ne laissera pas de la place à tout le monde, à tous les satellites et systèmes spatiaux placés en orbite. Il y aura donc une compétition croissante.

et à agir avant qu'il ne soit définitivement trop tard.

le passage d'une activité spatiale militaire purement stratégique à un usage plus lié aux opérations elles-mêmes- la guerre en Ukraine a démontré l'accélération de l'utilisation des données spatiales en soutien des opérations de combat deuxièmement, la multiplication du nombre de satellites en orbite ; troisièmement, une « arsenalisation » de l'espace, qui transforme les satellites en cibles potentielles. Par exemple, en 2019 et 2021, l'Inde, puis la Russie ont procédé à des tests antisatellites destructifs. En tant que puissance spatiale, la France a besoin de protéger ses matériels et, plus largement, ses intérêts. Sa capacité d'action dépend de son aptitude à surveiller l'environnement spatial pour détecter, puis attribuer les actes inamicaux

concerne l'amendement n° 133, on peut regretter, avec Pierre Laurent, que l'espace soit devenu un champ de conflictualité, mais ne pas prendre en compte cette nouvelle donne risque de

a recueilli l'avis favorable de la commission, puisqu'il tend à préciser que les capacités spatiales françaises futures devront être en mesure de détecter et d'attribuer les actions menées dans l'espace. On sait qu'il y a déjà eu un certain nombre d'incidents et cette recommandation est utile. monsieur le ministre,

phrases y fait référence : « La stratégie spatiale de défense sera actualisée afin de prendre en compte des enjeux opérationnels de la très haute altitude. » Il faut un peu plus

un haut niveau d'ambition. L'objet de cet amendement est donc de préciser ce que doivent être ces ambitions stratégiques majeures, en évitant de réduire les intérêts français à ses seuls satellites militaires et en impliquant nos partenaires alliés,

L'espace est de plus en plus encombré par ce qu'on appelle les débris spatiaux, objets fabriqués par l'homme et lancés dans l'espace qui, au fil du temps, se désintègrent et forment des débris. Il peut s'agir de restes de satellites, de morceaux de lanceurs ou de fragments issus de la collision entre deux objets plus volumineux. Le problème est que l'on constate une prolifération exponentielle de ces débris dans l'espace. Aujourd'hui, quatre pays développent des missiles antisatellites : les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. Outre qu'ils sont inutiles, les missiles de ce genre produisent une quantité monstre de mini-débris spatiaux. Ces débris spatiaux sont source de dangerosité, car ils se déplacent en nuages à des vitesses hypersoniques, ce qui peut causer des dégâts à d'autres satellites et, ainsi, produire de nouveaux débris. C'est le syndrome de Kessler, du nom de l'astrophysicien qui a théorisé ce phénomène : deux débris qui entrent en collision génèrent une profusion de débris, qui, à leur tour, vont engendrer de nouvelles collisions et de nouveaux débris. La Station spatiale internationale (ISS) doit régulièrement modifier son orbite pour éviter des débris spatiaux. Si elle est touchée, son intégrité structurelle sera sérieusement affectée, ce qui mènera à sa désintégration.

de débris spatiaux, particulièrement à longue durée de vie ». Nous nous inscrivons dans un souci de sécurité spatiale. Nous souhaitons également que la recherche militaire visant notre développement capacitaire dans l'espace étudie les moyens de collecter ces déchets pour améliorer là aussi la sécurité spatiale.

Par ailleurs, la France applique scrupuleusement les recommandations du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de l'ONU, qui invite déjà, depuis un certain temps, à « éviter la destruction intentionnelle de tout engin spatial ». Avis défavorable.

Gréaume. Cet amendement vise à promouvoir une réelle diversification de nos partenariats stratégiques afin de tisser des alliances en fonction des intérêts propres à notre nation, et non à ceux du bloc atlantiste et,, des États-Unis. La France, dans son propre intérêt, doit venir en appui aux pays, de plus en plus nombreux, qui refusent l'alignement derrière la Russie, mais aussi derrière l'Otan, et qui se donnent pour but la construction commune de la paix par la sécurité collective et la poursuite d'objectifs partagés en matière de sécurité humaine, alimentaire, sanitaire, énergétique et climatique.

n'est pas véritablement problématique : la diversification des partenariats stratégiques, c'est déjà ce que la France pratique ! En revanche, s'il s'agit de substituer cette rédaction à la référence à nos partenariats stratégiques actuels, à nos alliés

Son trafic maritime est important pour nous. Elle constitue une voie majeure d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne et un formidable réservoir de la biodiversité. Malheureusement, depuis quelques années, elle est aussi devenue la route migratoire la plus meurtrière au monde. En ce qui concerne le elle est également une zone géographique critique, car disputée, avec un renforcement de la présence militaire de nombreux pays et le risque d'une escalade des tensions. Je crois que, si la France veut jouer un rôle stabilisateur, la trajectoire de renforcement de nos forces armées dans cette région doit être soutenue. C'est l'objet du

héritage lourd à porter. Elle a signé une douzaine d'accords de défense avec les pays d'Afrique francophone entre 1960 et 1963 et a conduit 52 interventions militaires en Afrique de 1964 à 2014.

Lecointre : « Je décrirai notre vision de l'approche globale comme une stratégie de gestion de crise centrée sur la population et sur sa perception du développement de la crise. Ce concept est hérité de notre aventure coloniale. »

Quel est l'avis de la commission ? La mention de l'ancien empire colonial français relève d'une prise de position politique que ne partage pas la commission. Avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Défavorable.

des fins d'analyse, de compréhension et d'échange de bonnes pratiques avec les armées partenaires.

notamment sur le développement des bases françaises. Dans son discours du 27 février dernier, le Président de la République a annoncé l'allégement de notre présence militaire en Afrique et son redéploiement. Cet amendement vise à souligner le fait que l'implantation ou le maintien de chacune de nos bases doit se faire avec

le maintien d'une présence militaire française. Je ne vois pas au nom de quoi nous les abandonnerions, surtout au moment où dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le risque et la pression terroristes sont malheureusement en train de renaître.

Elles le sont aussi pour la préservation des intérêts de la France et pour la protection de nos ressortissants. Ainsi, l'opération Sagittaire, qui a été menée de main de maître par nos militaires, n'aurait peut-être pas pu avoir

croyez-moi -à ne plus vouloir porter d'étiquette politico-militaire avant de se rendre dans des zones de conflit extrêmement dangereuses pour y apporter de l'aide alimentaire

nous soutenons cette stratégie, même si la commission a pointé à de nombreuses reprises ses difficultés et ses insuffisances. Bien évidemment, pour pouvoir mettre en oeuvre un peu de diplomatie et beaucoup de développement, il faut parfois l'intervention de la défense afin de sécuriser les zones.

En ce sens, nous souhaitons que, parallèlement à son effort de défense, la France fasse de nouveau vivre les idéaux de paix, seuls à même d'éviter un conflit mondial généralisé.

Monsieur le ministre,

Mme Michelle Gréaume. Le rattrapage du point d'indice est un combat commun à tous les fonctionnaires. La dernière annonce de revalorisation faite par le ministre Guerini s'est avérée largement insuffisante et le contexte inflationniste place les agents de la défense dans une attente forte. Je tiens d'ailleurs à rappeler que ce contexte inflationniste n'a pas débuté avec la guerre en Ukraine, mais à la fin du premier semestre de 2021. Remplir le réfrigérateur, accéder aux loisirs et à la culture, partir en vacances, tout cela devient de plus en plus difficile pour bon nombre de travailleurs.

C'est pourquoi, à travers cet amendement, nous demandons une réforme du point d'indice pour procéder notamment à son dégel. Selon le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), les militaires souhaiteraient même un choc indiciaire. Je vous prie, monsieur le ministre, d'entendre leur voix. Quel

dans le détail, les femmes représentent 61,2 % des effectifs du service de santé, 31,6 % des personnels du commissariat des armées, 23 % des effectifs de l'armée de l'air, 15,2 % des effectifs de la marine nationale, et seulement 11 % des effectifs de l'armée de terre. Le plafond de verre et la discrimination qui subsistent ne sont pas acceptables. Il n'existe en effet aucune raison valable de ne pas reconnaître et de ne pas valoriser les compétences, les talents et les perspectives de carrière des femmes, au même titre que ceux de leurs homologues masculins.

aux générations futures et encourage les jeunes femmes à envisager des carrières militaires et à exercer des postes à responsabilité. Il démontre également que les femmes peuvent occuper des postes de pouvoir et d'autorité au sein de ces institutions.

est ainsi libellé : La parole est à M. Daniel Salmon. Par cet amendement, nous demandons la mise en place d'une journée de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu'à toute forme de discrimination dans les écoles qui dépendent du ministère des armées.

C'est ainsi que des comportements misogynes, LGBTQI+phobes ou racistes tendent à persister. Quant aux violences sexistes et sexuelles, une enquête interne de l'École polytechnique menée l'année dernière montre l'ampleur du phénomène 23 % des étudiantes affirment avoir été victimes d'une agression sexuelle pendant leur scolarité ; onze personnes ont été victimes de viol ou de tentative de viol. Pour sortir de ce climat que l'on peut qualifier d'infernal et pour mettre fin à ces pratiques, nous proposons la mise en place d'une journée de sensibilisation, à l'image de la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme.

le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l'insertion professionnelle des conjoints des militaires et sur les mesures d'accompagnement que le Gouvernement met en place pour leurs carrières professionnelles. D'une certaine façon, madame la

En effet, comment servir dans une armée, si l'on est trop souvent confronté à des remarques misogynes ou homophobes ? Comment servir dans une armée, si le harcèlement est quasi quotidien ? C'est évidemment impossible. Nous devons renforcer la lutte contre les discriminations et le harcèlement dans l'armée. C'est la raison pour laquelle, nous proposons, d'une part, de rappeler cet impératif de lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexuelles et sexistes, ainsi que celles qui sont liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre et, d'autre part, de modifier le fonctionnement de la cellule Thémis, mise en place en 2014 pour traiter les signalements concernant les militaires. À l'heure actuelle, c'est généralement le supérieur ou la supérieure hiérarchique qui mène l'enquête après la saisine de la cellule. Or ce mode de fonctionnement ne permet pas de garantir l'indépendance des enquêtes, les supérieurs risquant de couvrir les auteurs des infractions.

de loi de programmation militaire présente une nouvelle fois la dissuasion nucléaire comme la clé de voûte de notre stratégie, mais il occulte complètement les très nombreuses victimes qui ont permis à l'État français de se doter d'un tel arsenal. Il est primordial que ces victimes puissent être indemnisées à la hauteur des préjudices

l'objectif de disposer de dix patrouilleurs hauturiers basés en métropole. Je rappelle que ces bâtiments ont vocation à remplacer les patrouilleurs de haute mer et les patrouilleurs de service public, qui effectuent de nombreuses missions et veillent à la sûreté de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.

Monsieur le président Cambon,

point à la ligne ! Et vous ne voulez pas l'entendre.

Merci, monsieur le président.

Monsieur le ministre, nous formons notre jugement en conscience. Nous avons écouté les arguments de la commission. Nous avons écouté vos réponses et je dois dire que vous ne m'avez pas convaincu. Vous avez défendu la politique de la solution unique. Vous avez utilisé des arguments d'autorité : vos services ont bien travaillé, je n'en doute pas.

en rien derrière un argument d'autorité. Je vous expose les ingrédients de la programmation : j'aimerais comprendre ceux que retient le Sénat, ce qui me permettra de me rapprocher de lui, non pas avec autorité, mais avec affection.